La séance est ouverte.. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 25 janvier 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été publiée.

que j'ai déposée, avec les présidents Bas et Retailleau, sur le développement durable des territoires littoraux, un texte qui me tient particulièrement à coeur et qui constitue même- je pèse mes mots -le sujet majeur de mon engagement de sénateur depuis mon élection, en 2014.

l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », du 3 janvier 1986. Il s'agit d'élus des départements littoraux, mais aussi de départements ayant des communes riveraines de lacs de plus de 1 000 hectares auxquelles la loi Littoral s'applique.

L'insécurité juridique est grande. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le législateur, avec l'appui du Gouvernement, doit clarifier et préciser les incertitudes et les excès de la jurisprudence. Je précise tout de suite, et avec force, que je suis particulièrement attaché à la loi Littoral, à son respect, à son esprit. Ce qui semble évident va sans doute mieux en le disant, tant sur ce sujet sensible la caricature est facile et le malentendu possiblement durable. Je suis attaché à la loi Littoral, comme le sont tous les élus locaux, très attentifs au débat qui se tient aujourd'hui en séance publique, qui se sont mobilisés au fil des années et des contentieux, et se sont structurés au sein de l'Association des maires de France, de l'Association nationale des élus du littoral, l'ANEL, que préside notre collègue Jean-François Rapin, ou encore au sein de l'Association des maires ruraux de France, l'AMRF, lesquelles soutiennent ce texte. Je ne manque pas de citer aussi les associations de particuliers créées par des propriétaires de biens immobiliers en zone littorale, comme les PLUmés, infatigables promoteurs d'une clarification législative des lois Littoral et ALUR. Il est peu de dire que tous sont extrêmement attentifs à l'examen et au devenir du texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui,

Quelques mots de la genèse de cette proposition de loi : à la fin de 2016 est parvenue au Sénat une proposition de loi déposée par des députés socialistes portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique et discutée à l'Assemblée au cours des semaines précédentes. Cette proposition de loi visait essentiellement à donner des outils aux élus locaux pour le redéploiement des activités lié au recul du trait de côte du fait de l'érosion, elle était d'ailleurs rapportée à l'Assemblée nationale par la députée de Gironde Pascale Got, qui avait dans sa circonscription la commune de Soulac-sur-Mer ainsi que l'immeuble Le Signal, particulièrement touchés par l'érosion. Rapporteur du texte transmis au Sénat, j'avais souhaité conserver, bien sûr, le dispositif visant à lutter contre l'érosion du trait de côte, avec toutefois quelques réserves, notamment sur le fonds mis et apporter quelques aménagements supplémentaires pour régler les problèmes liés aux fluctuations jurisprudentielles autour de la loi Littoral. La commission de l'aménagement du territoire a voté ces aménagements et le texte ainsi amendé était largement adopté en séance en janvier 2017. nationale a ensuite examiné le texte en seconde lecture un mois plus tard, avant que la séquence électorale n'intervienne et ne précipite l'agenda parlementaire. Le texte ne connut pas de seconde lecture au Sénat. À l'été 2017, j'ai repris dans un nouveau texte les grandes lignes de la proposition de loi telle qu'elle résultait des travaux du Sénat, gardant le dispositif relatif au trait de côte, supprimant le dispositif, sensible et polémique, qui permettait d'aménager des zones d'activités en discontinuité de l'urbanisation existante. Avec l'appui majeur des présidents Retailleau et Bas, j'ai ainsi déposé la proposition de loi soumise à notre examen aujourd'hui, permettant ainsi au nouveau gouvernement et à la nouvelle majorité de prendre le temps de l'étude et de la réflexion. Avec le rapporteur Didier Mandelli, élu de Vendée dont l'implication est totale, nous avons mené de très nombreuses auditions, à Paris, dans le Finistère, en Vendée, qui confortent et consolident le texte, et ont aussi conduit à quelques aménagements de précision. De façon centrale, le texte réécrit prévoit l'urbanisation des « dents creuses » dans les hameaux et villages, l'accès à la mer pour les professionnels et la possibilité de construire des abris de jardins et annexes, avec des clauses interdisant le changement d'affectation. J'espère

en évitant toutes les caricatures, qui ne seraient pas à la hauteur du débat attendu par nos collègues élus et de l'engagement du Président de la République lors du Congrès des maires, que je veux ici citer Qu'y a-t-il de commun entre un centre-bourg, une métropole, une commune qui relève de la loi Montagne ou celle qui relève tout entière de la loi Littoral de manière parfois totalement inadaptée ? Des rigidités pensées pour parfois toute une catégorie alors que ça ne correspond pas à la réalité locale ! Des spécificités qui parfois créent d'autres contraintes, cela aussi, nous devons le changer. »

-, l'urbanisation doit être possible dès lors qu'il y a un petit ensemble de maisons d'habitation- cinq à huit maisons serait sûrement le bon seuil. De même, la définition d'une dent creuse doit être trouvée. Dans notre esprit, une parcelle insérée dans un ensemble construit est une dent creuse. insérée dans un ensemble construit est une dent creuse. Cela va dans le sens de l'économie du foncier et d'une meilleure préservation des terres agricoles. Très bien ! Si nous nous en tenons au texte, ce dispositif ne peut être

L'accès des professionnels à la mer peut permettre le développement d'activités telles que les cultures marines, la conchyliculture et les aménagements publics liés à la mer dans les espaces proches du rivage. Enfin, le texte prévoit la possibilité, comme ce fut le cas avec la loi Montagne votée en 2016, de construire des abris de jardins et des annexes de dimensions limitées sans possibilité de changement d'affectation. Le législateur a le devoir de s'emparer de ce sujet, même s'il est difficile. C'est indispensable si nous voulons éviter que, du fait de l'insécurité juridique, de nombreuses communes soient condamnées à verser de fortes indemnités des autorisations, ou opposé des refus, de certificat d'urbanisme ou de permis de construire, et si nous ne souhaitons pas refermer de façon excessive les possibilités d'évolution de nos communes littorales.

J'ai donc confiance, puisque la volonté exprimée par votre mouvement est d'apporter des solutions concrètes aux difficultés et aux blocages, de respecter les engagements pris- je pense, bien sûr, à celui du Président de la République sur le sujet lors du Congrès des maires. Enfin, je ne doute pas que vous et votre mouvement, qui êtes attentifs à préférer l'intérêt général à toute position partisane, aurez à coeur, après la première lecture au Sénat, de faire en sorte que ce texte puisse poursuivre son cheminement législatif dans le respect de nos institutions démocratiques et de leur pluralité.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, déposée le 13 septembre 2017 par Michel Vaspart, dont je salue l'opiniâtreté, ... Il a raison ! ... Bruno Retailleau, Philippe Bas et nombre de nos collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste. Ce texte vise à relancer le processus d'examen des dispositions de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, que le Sénat avait adoptée le 11 janvier 2017 en première lecture. Toutefois, l'examen de ce texte avait été interrompu par la suspension des travaux parlementaires préalable aux élections. La présente proposition de loi reprend donc fidèlement le précédent texte tel qu'adopté par le Sénat en première lecture. À cet égard, je tiens à saluer l'excellent travail mené à l'époque par nos collègues Michel Vaspart, rapporteur de notre commission, et Philippe Bas, président et rapporteur pour avis de la commission des lois, qui s'est à nouveau saisie pour avis. Le principal objectif du texte est de mieux prendre en compte le phénomène du recul du trait de côte dans les politiques d'aménagement. Je rappelle que le trait de côte représente environ 5 800 kilomètres pour la France métropolitaine et près de 10 000 kilomètres pour les outre-mer, l'on estime qu'un quart de la côte- environ 22 %-connaît un phénomène d'érosion marquée, auquel s'ajoute l'élévation du niveau de la mer, accélérée par le changement climatique. La gravité de certaines situations, dont est emblématique l'immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer, en Gironde, appelle une réponse rapide de la part des pouvoirs publics, pour les résoudre dans des conditions équitables, mais aussi pour éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir. Il nous faut donc développer un aménagement du territoire véritablement prospectif pour concilier l'incertitude et la précarité qui résultent du recul du trait de côte, avec le maintien d'activités dans les espaces concernés. Pour cela, le texte prévoit la mise en place d'une série d'instruments nouveaux. Il crée ainsi des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, des zones d'activité résiliente et temporaire, ou ZART, un nouveau bail réel immobilier littoral, ou BRILi, et la possibilité de mobiliser le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, également appelé « fonds Barnier », pour financer certaines opérations d'aménagement. Comme ce point a été évoqué lors de nos auditions, je précise qu'une meilleure prise en compte du recul du trait de côte dans l'aménagement du littoral n'implique aucunement de renoncer à lutter par ailleurs contre ce phénomène, par des ouvrages de défense contre la mer qui soient à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas l'objet du texte, mais c'est un sujet qui en est indissociable, madame la secrétaire d'État, et pour lequel nous souhaitons une présence et un soutien forts de l'État, car il s'agit d'une mission véritablement régalienne de protection des des populations et des biens. Permettez-moi, par ailleurs, de déplorer à nouveau le plafonnement des recettes du fonds Barnier à 137 millions d'euros par la loi de finances pour 2018, qui contraint durablement ses capacités d'intervention. Dans sa grande sagesse, le Sénat avait supprimé ce plafond, qui a été finalement rétabli en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Dommage ! Le texte que nous examinons reprend également un ajout du Sénat dans la précédente proposition de loi permettant de déroger au principe d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante dans les communes littorales, pour certaines opérations. L'article 9 vise ainsi la densification des hameaux, la relocalisation de constructions dans le cadre d'une ZART, les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines, et l'établissement d'annexes de taille limitée. de la précédente proposition de loi, cet article avait soulevé des réactions disproportionnées par rapport à la réalité du texte. En effet, les opérations visées sont strictement encadrées. Tout d'abord, elles ne peuvent pas cibler les espaces proches du rivage. Par ailleurs, elles doivent faire l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et elles ne peuvent être autorisées si elles portent atteinte à l'environnement ou aux paysages. Enfin, elles n'ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Ces nombreux garde-fous sont des forces de rappel considérables, qui permettront de prévenir les dérives. Tous les parlementaires ici présents partagent le souhait de voir préservé le patrimoine exceptionnel de nos territoires littoraux. Il nous semble néanmoins indispensable de faire évoluer l'état du droit, car les difficultés dans les territoires littoraux sont réelles, nombreuses, et durent depuis trop longtemps. Je rappelle que plus de 1 200 communes sont soumises au régime de la loi Littoral, sur l'ensemble de leur territoire, y compris les zones rétro-littorales éloignées du rivage. Notre commission avait adopté en 2014 un rapport très complet sur l'application de la loi Littoral, présenté par nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet. Ce travail a établi un constat clair, équilibré et transpartisan sur les difficultés rencontrées dans les territoires littoraux, qui a directement nourri le texte que nous examinons aujourd'hui. Constatant que le texte reprenait celui adopté par le Sénat il y a tout juste un an, notre commission a adopté des ajustements et des précisions en vue de conforter les orientations retenues. Sur plusieurs articles, nous avons mené ce travail en étroite collaboration avec le rapporteur pour avis de la commission des lois, poursuivant ainsi le travail mené lors du précédent texte, et je m'en félicite. Ainsi, la commission a supprimé l'article 6 prévoyant la transmission par l'État aux collectivités territoriales d'un document unique relatif aux risques naturels existant sur leur territoire, considérant que cette disposition pouvait être source de complexité et de rigidité, dès lors que le « porter à connaissance » s'effectue aujourd'hui en continu. Jugeant que la rédaction proposée à l'article 9 offre un équilibre entre les impératifs de protection et d'aménagement du littoral, la commission n'a pas jugé opportun d'infléchir significativement son contenu. Elle n'a procédé qu'à un ajustement relatif aux cultures marines, avec un accès direct à la mer, comme le souhaitaient les professionnels. Elle a par ailleurs réécrit l'article 12 relatif à l'intégration des risques naturels dans l'évaluation environnementale des projets, en privilégiant un enrichissement de l'étude d'impact. La commission a également souhaité sécuriser plusieurs outils mis à disposition des collectivités : les opérations d'aménagement dans les ZART prévues à l'article 15, le contrat de bail réel immobilier littoral, le BRILi, institué à l'article 16, et la mobilisation du fonds Barnier pour financer l'adaptation au recul du trait de côte,

Qu'y a-t-il de commun entre un centre-bourg, une métropole, une commune qui relève de la loi Montagne ou celle qui relève tout entière de la loi Littoral de manière parfois totalement inadaptée ? Des rigidités pensées pour parfois toute une catégorie alors que ça ne correspond pas à la réalité locale ! Plutôt que d'avoir des débats théoriques pour savoir comment on traite tout le pays de la même façon, ayons une approche pragmatique, différenciée. Permettons de faire. Laissons les maires innover.

et de l'existant, en vue de mieux tenir compte des spécificités locales et de l'histoire vécue depuis 1986 par toutes les collectivités locales. Sur ces Sur ces sujets, l'inaction n'est plus une option. Les enjeux liés au recul du trait de côte sont trop urgents et les problématiques relatives à l'urbanisation sont trop anciennes pour remettre sans cesse à plus tard la recherche de solutions. Notre objectif est de retrouver l'esprit de la loi Littoral, par une application pleine et entière du principe de développement durable de tous ces territoires. La parole est à M. le rapporteur

et des mesures ponctuelles, limitées, parfaitement circonscrites, permettant, sans porter atteinte aux principes de la loi Littoral, de faciliter des constructions en dehors du rivage, sans vue sur la mer et sur autorisation du préfet, uniquement dans des hameaux, qu'il ne s'agit pas d'étendre, mais à l'intérieur desquels il y a déjà des constructions et, entre ces constructions, des terrains à bâtir.

Au contraire, nous en mesurons tout l'apport pour défendre une richesse essentielle qui, dans un département comme le mien, la Manche, a été parfaitement préservée. Les bétonneurs ne sont pas chez nous et ils ont, heureusement, été arrêtés par la loi Littoral, laquelle a joué un rôle historique indispensable

ont cherché à combler, non pas des dents creuses, mais des vides juridiques. La loi Littoral, elle-même, est très générale. Des juridictions, même en l'absence d'inconvénients pour la protection du littoral, ont interdit de construire sur des terrains appartenant à des propriétaires privés, lesquels sont souvent des personnes qui attendent l'approche de la retraite pour faire construire,

Il s'agit spécifiquement de ces cas tout à fait particuliers, pour lesquels nous souhaitons apporter une solution parfaitement pragmatique, et en mettant en place des garanties fondamentales. Premièrement, aucune construction n'est possible

et l'on ne voit pas comment elles pourraient être transgressées au point de menacer le moins du monde la protection du littoral. Voilà pourquoi, madame la secrétaire d'État, j'attends avec confiance d'entendre le propos que vous tiendrez à la tribune.

mer. Il est plus que jamais impératif de repenser l'élaboration de nos politiques publiques et d'anticiper les effets du changement climatique pour imaginer, penser le littoral de demain

12 % de la population française. Entre 2000 et 2006, l'artificialisation des sols y était encore près de trois fois plus élevée que la moyenne nationale.

raison pour laquelle, dans ce contexte, le Gouvernement salue votre initiative. S'agissant de ces phénomènes d'érosion et de gestion du trait de côte, deux questions principales nous semblent en effet devoir être rapidement traitées.

On sait que l'organisation du repli des activités concernées est absolument primordiale- je l'ai évoquée avec certains d'entre vous ces derniers jours. Cela signifie que la relocalisation de certaines activités, de certains quartiers, voire, à plus long terme, de villes entières, à l'intérieur des terres

il faut aborder la question, déjà d'actualité, du financement des opérations de relocalisation ou d'indemnisation des biens concernés par le recul côtier. Tels sont les deux aspects qui nous paraissent essentiels et qui structurent notre approche. Votre texte, messieurs les sénateurs, pose donc la question des modalités de prise en compte du recul côtier. La spécificité du phénomène d'érosion appelle des solutions nouvelles qui privilégient l'anticipation et l'adaptation. Ce phénomène intéresse tout d'abord, et en premier chef, les territoires et leur aménagement dans toutes leurs spécificités. fin, il faut améliorer les outils des collectivités compétentes en matière d'aménagement du territoire et faire évoluer le cadre juridique existant pour permettre aux territoires concernés de bien prendre en compte la temporalité de ce phénomène dans leurs documents d'urbanisme.

: il faut garder en mémoire et à l'esprit le fait qu'une dune ou une mangrove préservée constitue un des remparts les plus efficaces et les moins coûteux contre la subversion marine.

Les orientations que je viens d'énumérer vont à l'encontre de la logique de gestion des risques qui prévaut dans la proposition de loi. L'approche des plans de prévention nous semble mal adaptée au regard de la spécificité du phénomène évoqué. la réalisation de plans intégrant l'érosion du trait de côte a pu parfois apporter une première réponse dans certains territoires. En revanche, cela a conduit à interdire toute construction dans la zone impactée par l'érosion à un horizon de cent ans. Or, s'il est pertinent d'interdire des constructions dans des zones soumises à des risques pouvant se produire à tout moment, il paraît disproportionné de « geler » des territoires qui seront atteints par l'érosion à un horizon parfois éloigné, mais toujours prévisible. C'est la caractéristique de l'évolution du trait de côte. Au-delà, il apparaît également nécessaire, à nos yeux, de bien informer la population, notamment les acquéreurs de biens exposés à l'érosion, et de responsabiliser les constructeurs de bâtiments nouveaux.

doivent être trouvées, et nous allons y travailler. L'État doit être en mesure d'accompagner certaines expérimentations, ... Il y a urgence ! ... mais, en tout état de cause, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs ne peut pas être mobilisé pour ces opérations.

Ensuite, il y a la question de l'indemnisation des biens atteints par l'érosion tant que les projets d'adaptation précédemment évoqués ne seront pas mis en oeuvre. Cette question d'actualité fait débat. C'est notamment le cas de l'immeuble Le Signal en Gironde- vous le connaissez tous-, qui a d'ailleurs fortement influencé le contenu et l'orientation de la proposition de loi déposée dans le cadre de la précédente législature par Mmes Got et Berthelot. Votre proposition de loi, qui mobilise la solidarité nationale pour une indemnisation à 100 % ne s'inscrit pas dans la logique que souhaite développer le Gouvernement. Aucun des dispositifs actuels ne permet d'ailleurs de répondre pleinement aux enjeux de l'érosion côtière. Le Gouvernement travaille en conséquence à des propositions sur ce point afin de mettre en place rapidement un dispositif équitable et durable.

loi. Celle-ci date, certes, de 1986, mais elle a posé le principe de la préservation de nos côtes, qui font la richesse de nos territoires et l'identité de la France, face à une pression démographique et urbanistique qui continue

la loi Littoral demeure un pilier de la protection des espaces naturels littoraux et de la lutte contre l'artificialisation du territoire qu'il faut conforter. C'est vrai ! Nous que les débats relatifs à la question des principes de l'érosion côtière n'ont pas vocation, à ce stade, à porter sur l'évolution de certains des principes posés par la loi Littoral.

Cela dit, et je sais que nous en aurons l'occasion, nous pourrons travailler ensemble à l'avenir pour élaborer une proposition ou un projet de loi qui pourra aboutir. S'agissant des enjeux cruciaux de gestion de notre trait de côte, je crois nécessaire de promouvoir un dispositif plus intégré, comme le préconise notre stratégie nationale conciliant plusieurs politiques publiques et faisant appel à une pluralité d'acteurs.

-de solutions financières adaptées, notamment en ce qui concerne la question de l'indemnisation des biens menacés directement ou indirectement par l'érosion du trait de côte.

Les 27 juin et 1 juillet 1846, s'exprimant à la tribune de la chambre des pairs, Victor Hugo constatait la « dégradation de nos dunes et de nos falaises » et les « phénomènes qui menacent de ruiner une partie de nos ports et de déformer la configuration des côtes de France Ces propos sont toujours d'actualité et la question du trait de côte ainsi que le maintien et le développement d'activités sur le littoral sont au coeur du texte que nous examinons ce jour. Vous le savez, le trait de côte, selon le service hydrographique et océanographique de la marine,

Il est défini comme « la ligne portée sur la carte séparant la terre et la mer. Sur la carte marine, c'est le plus souvent la laisse de haute mer [c'est-à-dire] la ligne mince et ondulée formée de sable fin, de débris de coquilles, de petits morceaux d'algues, etc. laissée par les vagues, qui marque la limite supérieure atteinte par leur mouvement sur la plage. Le trait de côte connaît des mouvements d'ampleur, plus importants dans la période récente, comme l'a rappelé Mme la secrétaire d'État. Le Bureau de recherches géologiques et minières prévoit en effet une accélération de l'érosion et les chiffres sont clairs, voire alarmants. Les données que nous possédons sont plus inquiétantes que toutes les prédictions établies jusque-là. En 2025, le trait de côte devrait avoir reculé de 20 mètres sur la côte sableuse et de 9 mètres sur la côte rocheuse. En 2050, c'est pire et sans surprise : le recul serait de 50 mètres sur la côte sableuse et de 25 mètres sur la côte rocheuse. Au-delà du patrimoine que représente le littoral français, et du risque que fait peser sur celui-ci le recul du trait de côte, c'est surtout sur la grande diversité des situations qu'il convient d'insister. Le recul du trait de côte n'est pas uniforme, il n'a pas les mêmes incidences en baie de Somme, sur les falaises crayeuses de Normandie, les dunes d'Aquitaine ou dans les mangroves des territoires ultramarins. Seul un cadre juridique spécifique et suffisamment souple pourra être adapté à un problème qui, s'il ne se pose pas partout avec la même intensité ou les mêmes conséquences, est cependant généralisé, atteint des zones d'habitation ou d'activités, notamment saisonnières, de manière désormais parfaitement identifiée par les travaux scientifiques. Ce débat n'est pas nouveau et le Parlement s'en est emparé en 2017 avec une proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, débat qui avait été interrompu par la suspension des travaux parlementaires. Pour rafraîchir les mémoires, voilà ce que déclarait d'ailleurs la députée Pascale Got à l'occasion de la seconde lecture de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, en 2017, avant l'interruption du processus législatif : « Chers collègues, je vous demande d'arrêter le kidnapping de cette proposition de loi sur le recul du trait de côte. Je m'adresse à tous ceux qui se sont égarés, à tous ceux qui voudraient prendre, ce soir, le chemin de la déraison emprunté par certains sénateurs pour détricoter la loi Littoral : vous vous trompez de texte. » L'objet de ce courroux était le détricotage de la loi Littoral proposé par les sénateurs et que l'on retrouve une nouvelle fois dans cette proposition de loi, notamment dans son article 9. Nous entendons et admettons parfaitement que ce texte n'a pas pour seul objet de résoudre des situations ponctuelles, comme celle de l'immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer, sur laquelle porte l'article 3, même s'il convient d'élaborer d'urgence une solution applicable sans délai. Néanmoins, nous pensons que cette situation, toute particulière en raison de la nature de la construction sur une dune elle-même mouvante, ne nécessite pas d'être inscrite dans la loi et qu'il faut plutôt rechercher des solutions au cas par cas. Oui, nous partageons toutes et tous ici le sentiment qu'il est nécessaire de lever certains blocages dus à la loi Littoral, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quel cadre. S'il convient de trouver des moyens d'urbaniser nos côtes en ayant recours au sens commun,

L'article 9 n'aura d'autre finalité que de créer des contentieux, et chacun sait bien que les mauvais procès qui durent ne sont en rien un apport positif. La finalité du texte, pour ces auteurs, est de « mieux prendre en compte les effets du changement climatique en termes d'érosion et d'élévation du niveau de la mer, afin de concilier le risque de recul du trait de côte avec le maintien et le développement d'activités dans les territoires littoraux ». Nous pouvons entendre cet argument et nous dire que certains volets de la proposition de loi méritent un examen attentif et bienveillant, mais, ayons aussi à l'esprit, mes chers collègues, que les mots ont un sens et que parler de risque est une preuve de légèreté qui mérite d'être battue en brèche. Nous savons aujourd'hui que le risque est avéré et que nous devons parler de certitudes, même si certains de nos collègues considèrent que, si submersion marine il doit y avoir, ce n'est pas pour demain et qu'il sera temps, le moment venu, de regarder les choses et de prendre les mesures qui conviennent. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette vision et nous avons l'impérieux devoir d'imaginer, d'anticiper et de tenter d'éviter le pire. C'est bien le sens de l'action politique que de regarder la situation en face et non pas à l'aune de telle ou telle situation particulière. Certains me rétorqueront qu'en tant qu'élu de la métropole lilloise, je ne suis pas le plus habilité pour évoquer les questions relatives au littoral. Je viens d'une région, les Hauts-de-France, riche d'un littoral long de 190 kilomètres, soumis à de multiples défis, qu'il s'agisse des risques ponctuels comme les submersions marines ou de transformations plus structurelles résultant du recul du trait de côte. La philosophie générale de ce texte et ses attendus me conduisent à dire que cette proposition de loi est, au fond, une fausse bonne idée. Vous l'avez dit, madame la secrétaire d'État, le sujet mérite une réflexion collective associant la représentation nationale dans son ensemble et le Gouvernement, et non pas cette seule initiative. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche ne votera pas cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'objectif de cette proposition de loi- garantir de nouveaux instruments à l'État et aux élus locaux pour faire face au recul du trait de côte lié à l'érosion et à la montée des eaux

Nous sommes loin de la simplification des normes, objectif souvent affiché dans cette maison. Nous nous posons également des questions sur l'opérationnalité des mesures proposées.

Cela suppose des moyens d'expertise et des moyens financiers. Nous connaissons tous la situation actuelle des collectivités qui voient leurs dotations diminuer, loi de finances après loi de finances. Il est intéressant de donner des outils, mais encore faut-il avoir les moyens de s'en servir. Sur le fond, ce dispositif nous interroge : l'objectif n'est pas d'empêcher la construction ou le maintien de constructions, mais bien de créer les conditions de leur aménagement. Nous proposerons donc des garde-fous pour que ces nouvelles zones ne se situent pas dans les espaces les plus touchés par le risque de submersion, soit les anciennes zones rouges. Nous avons également des interrogations sur les nouvelles responsabilités confiées au fonds Barnier, dont les ressources diminuent progressivement. Cette année, la taxe affectée à ce fonds est plafonnée à hauteur de 137 millions d'euros, ce qui permet de reverser 90 millions d'euros au budget général. Ce montant est très inférieur aux dépenses constatées ces dernières années, équivalentes à 178 millions d'euros. Cette inquiétude est renforcée par la situation du budget consacré aux risques hydrauliques et naturels, en constante régression, et le manque d'aboutissement des plans de prévention des risques naturels Il est indispensable que l'État prenne ses responsabilités face aux risques de submersion liés à l'érosion des côtes et à la montée des eaux. Enfin, nous regrettons que la boîte de Pandore de la loi Littoral soit une nouvelle fois ouverte. Certes, cette loi a trente mais nous portons une conviction : la lutte contre le mitage en zone littorale reste une impérieuse nécessité. La protection des côtes et la préservation des terres agricoles ne peuvent être remises en cause. Le principe de l'urbanisation continue est intéressant, même si sa définition trop imprécise questionne. Avant de complexifier en ajoutant des exceptions aux exceptions, il aurait été plus juste de mener un travail de définition sur les notions qui conditionnent la possibilité de construction dans ces zones et qui sont l'objet d'une jurisprudence fournie. Aujourd'hui, le seul élément réglementaire existant est une instruction gouvernementale de 2015. Il est primordial que soient mieux précisées les notions d'agglomération, de village, de hameau. Il est nécessaire que cette notion de hameau- « secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs » -soit plus clairement définie, pour permettre, sous certaines conditions, leur densification notamment dans les dents creuses. La jurisprudence concernant la loi Montagne est plus claire sur ce sujet. Dans mon secteur, un groupement est constitué à partir de quatre maisons distantes de moins de 50 mètres. Une définition claire et précise permettrait de sécuriser les procédures et le choix des élus. Elle est également souhaitable pour éviter que le préfet ne se trouve dans une situation discrétionnaire au moment d'autoriser ou non des projets d'urbanisation au regard de critères aujourd'hui flous et évolutifs, définis exclusivement par la jurisprudence. Il existe aujourd'hui une contradiction : il est plus facile de créer de nouveaux foyers d'urbanisation les « hameaux nouveaux » plutôt que de densifier le bâti existant au sein des hameaux. C'est un problème qu'il est impératif de résoudre, mais certainement pas en permettant tout et n'importe quoi. En effet, l'article 9 pose une dérogation extrêmement large en rendant possible une densification des hameaux qui respecterait « les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ». Il n'est aucunement fait référence au caractère regroupé et structuré des habitations. La voie est donc ouverte à une urbanisation extensive. Cette dérogation ne se limite pas au comblement des dents creuses, c'est-à-dire la construction d'une parcelle située entre deux parcelles construites, mais risque bien d'ouvrir un véritable droit au mitage. Je n'évoquerai pas les autres dérogations auxquelles nous sommes évidemment défavorables, notamment concernant l'implantation de constructions ou d'installations agricoles, exceptions qui existent déjà aujourd'hui, mais strictement limitées aux installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Permettre de construire en discontinuité urbaine pour la relocalisation des constructions et ouvrages de la ZART est également dangereux, tout comme la construction d'annexes non mitoyennes. Nous proposerons donc une réécriture de cet article en supprimant la notion de « hameau nouveau » et en autorisant la construction extrêmement limitée et encadrée dans les dents creuses des hameaux. Nous renvoyons à un décret la définition des notions qui conditionnent l'urbanisation. Au final, il ne faut pas se tromper d'objectif. Il s'agit bien d'accompagner les territoires devant les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique qui modifient les conditions de vie autour du littoral, et non de faciliter l'urbanisation le long du littoral. En l'état, nous ne pouvons voter ce texte.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, c'est après une année complète que nous reprenons les discussions sur ce sujet particulièrement important pour les territoires littoraux. Je tiens avant tout à remercier mes collègues Michel Vaspart, Bruno Retailleau et Philippe Bas, à l'origine de l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de notre assemblée.

Ce texte poursuit un triple objectif, comme cela vient d'être rappelé : préserver le littoral d'un urbanisme inconséquent, apporter une réponse circonscrite à la constructibilité dans les hameaux et sécuriser les documents d'urbanisme délivrés par les élus. Si les attentes des élus sont fortes, les craintes ou plutôt les réticences le sont tout autant. Elles se sont d'ailleurs manifestées dès l'adoption du texte par le Sénat en février 2017 une pétition intitulée « Ne touchez pas à la loi Littoral » avait même récolté 300 000 signatures. Pour certains, en effet, le littoral doit être sanctuarisé et la loi Littoral ne doit pas être modifiée. Pour d'autres, la protection du littoral est certes une véritable priorité, mais qui ne doit pas pour autant empêcher de faire évoluer un régime juridique afin de l'adapter aux enjeux actuels. C'est le cas des membres du groupe Union Centriste et des auteurs de cette proposition de loi. Quels sont les enjeux de ce texte ? Nous sommes au coeur de l'hiver, en janvier, et déjà deux tempêtes majeures ont traversé notre pays en provoquant des dégâts parfois très importants. Le recul du trait de côte est l'une des conséquences de ces tempêtes, particulièrement visible sur les côtes sablonneuses. Il faut donc envisager non seulement de protéger les populations les plus directement concernées, c'est-à-dire celles dont les habitations menacent de s'effondrer, mais aussi anticiper en relocalisant les habitations et les activités économiques plus en amont. Cela implique de créer des outils ou d'adapter ceux qui existent afin de permettre aux pouvoirs publics- les élus locaux et les préfets -d'anticiper. Cette adaptation des outils d'urbanisme doit préserver l'équilibre trouvé par la loi Littoral afin de protéger nos côtes d'une « bétonisation » excessive. Il s'agit bien de trouver des dispositions équilibrées, entre la protection des populations et de l'environnement et la possibilité de maintenir des activités économiques sur le littoral. Parmi ces outils figurent les zones d'activité résiliente et temporaire, c'est-à-dire le maintien de constructions dans des zones qui pourraient être menacées par un recul du trait de côte, mais qui ne le sont pas dans l'immédiat. Cet outil apporte une souplesse supplémentaire bienvenue pour les professionnels dont l'activité impose un accès à la mer : conchyliculteurs, activités nautiques. Le Sénat avait veillé l'an dernier Le Sénat avait veillé l'an dernier à bien l'intégrer dans le corpus de règles existant, et à permettre aux élus locaux d'en avoir l'initiative. Ces outils seront très utiles en Vendée, par exemple, où les activités nécessitant une proximité de la mer sont nombreuses. Associée aux ZART, la création du bail réel immobilier littoral permettra aux collectivités de développer, si elles le souhaitent, les espaces soumis à un risque potentiel de recul du trait de côte. Les relations entre le bailleur et le preneur sont adaptées à ce risque, notamment s'agissant de la répartition des frais de démolition si le risque se réalise. Le dispositif, qui figurait dans la proposition initiale, est sécurisé du point de vue juridique. L'article 9 de la proposition de loi a fait l'objet de nombreuses discussions en commission, les positions s'étant d'ailleurs durcies par rapport à l'an dernier. Les dérogations apportées au principe d'extension en continuité de l'urbanisation dans les parties rétro-littorales des communes, introduites par la majorité sénatoriale, avaient été diversement accueillies. Elles ont donc été retirées de la version que nous examinons aujourd'hui. Je salue tout de même l'amendement du rapporteur qui vise à permettre aux installations et constructions liées aux cultures marines d'être autorisées dans les espaces proches du rivage. Enfin, parmi les dispositions contestées, demeurent les possibilités de relocalisation d'activités subissant le recul du trait de côte et les mesures de comblement des dents creuses des hameaux.

respect des proportions en hauteur et en volume du bâti existant -sont de nature à dissiper les craintes de voir le littoral se densifier outre mesure. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis particulièrement attachée à la loi Littoral. En vigueur depuis 1986, elle a protégé nos côtes d'une urbanisation irraisonnée, et nous permet aujourd'hui de nous prévaloir d'un patrimoine naturel exceptionnel. Il n'est nullement question de remettre en cause les protections mises en oeuvre par cette loi dont les élus du littoral sont si fiers et auxquelles ils sont si attachés. Pour autant, ne nous interdisons pas d'en revoir certaines dispositions pour les adapter à des enjeux qui n'étaient pas- ou mal -connus dans les années Le recul du trait de côte est une réalité, dont les effets vont s'accentuer. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. N'ayons pas une vision dogmatique, mais soyons pragmatiques. Il faut permettre aux activités économiques de ces territoires littoraux et à nos communes de vivre, car elles font également

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte important, qui reprend en quasi-totalité les dispositions de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, déposée à l'origine, voilà un an,

La proposition de loi socialiste initiale partait d'un constat double : d'une part, l'élévation du niveau des eaux et les risques qui y sont liés- la submersion marine ou les inondations -et, d'autre part, une activité humaine de plus en plus importante sur le littoral, avec une pression sur la construction de logements trois fois plus forte que la moyenne nationale. Il s'agit d'un texte essentiel, qui mérite toute notre attention, puisque l'érosion côtière affecte 25 % de notre territoire métropolitain. La France compte près de 19 200 kilomètres de littoral ; c'est un réel atout naturel et économique, mais cela nous oblige aussi à prendre nos responsabilités. La longueur du trait de côte, quant à lui, représente environ 8 600 de loi de 2017 visait à répondre, dans le cadre de la prévention du risque, « au besoin de préservation des espaces et de sécurisation des populations, tout en organisant les conditions du maintien du dynamisme et du développement durable de nos côtes Alors que s'est conclue à Paris, voilà un peu plus de deux ans, la plus grande conférence mondiale sur le climat, la réalité des conséquences de la déréglementation climatique s'impose aujourd'hui régulièrement à nous. Cela entraîne inéluctablement une érosion côtière vérifiable et le recul, de fait, du trait de côte. Par ailleurs, une activité humaine de plus en plus développée sur ces territoires fragilisés accentue les effets de ces événements déjà prégnants

dernier, plusieurs milliers de mètres cubes de roches se sont écroulés au Tréport. À chaque fois, ces éboulements représentent une menace pour les personnes et les biens, mais ils affectent également les activités touristiques. C'est la raison pour laquelle le phénomène d'érosion côtière ne peut plus donner lieu à des réactions laxistes, au prétexte que son effet est continu dans le temps et moins visible qu'une inondation. Les risques y afférents, qu'ils concernent les territoires, les biens ou les populations, sont réels et inquiétants, je viens de le souligner. Nous en avons désormais pleinement conscience, et il est de notre devoir d'anticiper les conséquences de cette évolution. C'est l'intérêt de cet outil législatif, qui remédie aux actions et aux décisions prises dans l'urgence, à la suite d'un aléa, et qui apporte une solution juridique, en particulier, aux aux élus confrontés aux questions de relocalisation. Plusieurs dispositions ont déjà été mises en oeuvre, au cours des dernières années, dans ce domaine, et les deux propositions de loi s'inscrivent dans la continuité de ces actions. Néanmoins, celle que nous examinons aujourd'hui comporte malheureusement plusieurs mesures faisant l'objet de divergences significatives, qui appellent tout particulièrement notre attention ; ce

creuses. Ce texte tend à assouplir cette loi, en introduisant plusieurs dérogations au principe d'extension en continuité de l'urbanisation dans les parties rétro-littorales des communes littorales. particulier, son article 9 reprend en grande partie la rédaction que la droite sénatoriale a défendue en 2017, et ce malgré le compromis trouvé, je le rappelle, avec les députés de l'ancienne majorité,

la possibilité d'identifier des espaces situés dans des ZART et destinés à l'accueil d'activités et de biens devant être relocalisés. En outre, la proposition de loi, qui- faut-il le rappeler ? -concerne non seulement la France continentale, mais aussi l'outre-mer, nous paraît ne pas prendre en compte les attentes et les spécificités de ces territoires, en supprimant, en particulier, les zones de mobilité du trait de côte, les ZMTC. Ce texte comporte donc des mesures qui remettent en cause des dispositifs essentiels de la loi Littoral ; or nous savons tous non seulement qu'elle est indispensable à la préservation des milieux naturels, mais encore qu'elle constitue la seule possibilité de prévenir les risques et de protéger les biens et les personnes.

l'idée que la France devait se doter d'une stratégie nationale, réunissant les collectivités et l'État, et d'une méthodologie de gestion du trait de côte, de recul stratégique et de défense contre la mer. À la suite des travaux de ce comité opérationnel, un groupe de travail, animé par le député de la Manche- déjà ce département ! -, Alain Cousin,

Ils ont été mis sur la table, on les a discutés, et l'on était bien content d'avoir quelque chose ... Il est vrai que le financement était réglé dans des conditions ne plaisant pas à tout le monde, mais il y avait un effort,

Ce rapide rappel de l'histoire des prévisions en la matière doit donc nous amener à beaucoup de prudence dans nos décisions, car nous ne pouvons pas ignorer que le consensus scientifique du rapport du GIEC, relu, comme toujours, par les États,

ans, c'est déjà beaucoup moins sûr ; à cent ans, nous n'en savons rien aujourd'hui ... Il faut donc se préparer à laisser à l'océan des territoires qu'il grignotera inéluctablement, à lui abandonner des constructions parfois anciennes, et à se doter d'outils

tout de même un peu le sentiment que les mesures techniques développées, notamment les fameuses ZART- on y reviendra au cours du débat -, retardent une gestion assumée de cette montée des eaux, au profit de certains bricolages peu durables.

dont nous discuterons tout à l'heure, qui pose la question essentielle, me semble-t-il, de la péréquation et de la solidarité nationale, est un élément important et intéressant de ce débat ; nous pouvons nous en saisir utilement. Néanmoins, la ZART,

eaux. Il ne s'agit pas non plus de ne rien faire ; nous sommes d'accord sur le fait que certaines activités doivent suivre le recul du trait de côte- l'ostréiculture, la restauration touristique, la plaisance. Il faut effectivement des dispositifs adaptés pour ces activités que nous connaissons et que nous pouvons lister, mais ce n'est pas ce que permet de faire la ZART, qui est beaucoup plus large et qui constitue, d'une certaine manière, un contournement de la loi Littoral, au nom du dérèglement climatique- lequel a bon dos dans cette affaire La ZART risque de conduire à un imbroglio général et je pense même que les rapporteurs de la proposition de loi initiale- Jérôme Bignon en rappelait l'histoire -en étaient un peu conscients, puisqu'ils ont ajouté un bricolage supplémentaire qui, à mon avis, restera dans les cours d'histoire du droit administratif, le bail

tous autour de la table pour construire ce consensus à partir des cas précis que l'on connaît. Que l'aéroport de Brest-Guipavas soit bridé par la loi Littoral, en soi, est une aberration, et je peux vous citer d'autres

fort de ses diversités, le patrimoine littoral et maritime de la France constitue un atout formidable, cela a été souligné à de nombreuses reprises cet après-midi. La Côte d'Albâtre, avec les célèbres falaises d'Étretat ou encore celles de Varengeville-sur-Mer surmontées du cimetière marin, compte ainsi des pépites inestimables.

La préservation du littoral est donc un impératif, mais sa protection ne doit pas se faire au détriment de sa valorisation. La sanctuarisation systématique des espaces littoraux et des espaces et milieux remarquables ne contribue pas forcément à leur préservation. La proposition de loi, très attendue, de notre collègue Michel Vaspart reprend une précédente proposition de loi, devenue caduque, tout en réintroduisant dans la protection du littoral une dose de souplesse, qui rend le principe de développement durable applicable au littoral. Cet objectif de développement durable impose d'abord d'adapter la protection aux projets de chaque territoire littoral, de manière pragmatique. Les maires sont soumis à la double contrainte du respect des règles d'urbanisme fixées par la loi et de la nécessaire valorisation économique de leur commune. Les projets économiques, notamment en milieu rural, s'appuient essentiellement sur le maintien de l'activité agricole et sur le développement d'une activité touristique complémentaire. complémentaire. Conformément au principe du développement durable, ces projets ne s'opposent pas à la protection de l'environnement, dès lors qu'ils sont maîtrisés. L'article 9 de la proposition de loi, qui facilite la mise en oeuvre de projets agricoles essentiels pour la préservation des espaces naturels, répond à cet objectif. Ainsi, l'élevage participe à la préservation des côtes, en limitant, grâce aux pâturages, le ruissellement. la protection des espaces naturels de nos côtes doit pouvoir être conciliée avec la valorisation du patrimoine architectural sur les sites littoraux remarquables, quand ces espaces naturels littoraux font l'objet d'une « Opération grand site ».

Pour la défense contre la mer, le flou persistant sur l'interprétation de la notion d'ouvrage concerné, notamment sur les épis, repousse les investissements liés à leur maintenance et accroît le risque de recul du trait de côte. Enfin, l'ampleur des actions de lutte contre le retrait du trait de côte impose de donner aux collectivités, notamment aux communes, des moyens financiers à la hauteur des coûts de ces travaux. travaux. Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », créé en 1995, est aujourd'hui fortement altéré. Non seulement son champ d'action a été largement étendu sans véritable cohérence, mais surtout ses financements ont été plafonnés pour participer au redressement des comptes de la Nation. essentiel pour financer les actions de prévention contre les atteintes de la nature sur nos côtes, doit être garanti et son accès doit être ouvert aux mesures de prévention prises par les collectivités qui agissent contre l'érosion des côtes.

Maire pendant quinze ans d'une commune du Pas-de-Calais très concernée par le sujet de l'érosion, président de l'Association nationale des élus du littoral depuis 2012, je m'étais réjoui de voir aboutir un travail de plusieurs années entre les élus et l'État. En effet, à chaque nouvelle tempête, tous les élus du littoral constatent les effets du changement climatique. Les événements climatiques ayant affecté notre pays- des ouragans Irma, José et Maria ayant touché les Antilles, à la rentrée 2017,

Je salue d'ailleurs la mise en place à l'Assemblée nationale d'une mission d'information sur la gestion des événements climatiques majeurs dans les zones littorales, présidée par Maïna Sage, députée de la Polynésie française. Par essence, le littoral est instable et toujours en évolution. Nous en avons, au quotidien, des illustrations concrètes, sur nos rivages, liées à l'attaque des vagues et à l'érosion éolienne. À ces phénomènes s'ajoutent les effets des ouvrages de défense contre la mer, qui, construits pour protéger les côtes, ont parfois entraîné le dégraissement ou l'engraissement des plages. Depuis la tragédie de la tempête Xynthia, un travail considérable a été accompli par les services de l'État et par les élus.

qu'il semble nécessaire de trouver des solutions juridiques pour régler les situations d'urgence, ce qui n'exclut pas de réfléchir à de nouvelles formes d'urbanisme pour l'avenir. était l'objet de la proposition de loi initiale : adapter le droit à un trait de côte perpétuellement en mouvement et aux événements météorologiques violents, toujours plus fréquents. L'interruption de la session parlementaire a suspendu l'examen de ce texte. Est-on pour autant reparti de zéro ? Je ne le crois pas. Les événements climatiques de 2017 ont donné raison aux parlementaires qui avaient bien vu l'urgence d'un tel texte. J'ai en tête les images impressionnantes de l'ouragan Irma et, plus modestement, celles qui furent prises au début de ce mois sur la plage de la commune de Merlimont, dont j'ai été le maire, qui perd chaque année des tonnes de sable à cause du vent et des houles de plus en plus fortes.

la définition du recul du trait de côte, la reconnaissance juridique de la stratégie nationale et des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, la création de zones d'activité résiliente et temporaire, associées au bail réel immobilier littoral. Toutes ces innovations législatives ont été reconnues comme correspondant à un réel besoin des élus du littoral. Je soutiendrai donc ces dispositions, qui apportent des outils supplémentaires aux élus littoraux. Les discussions de l'an dernier nous ont aussi rappelé le fort attachement des Français à la loi Littoral, garante de la protection de nos côtes. J'ai toujours défendu cette loi et, au moment de fêter ses trente-deux ans d'existence, je la défendrai encore et je veillerai à l'application équilibrée de ses deux volets, préservation et développement du littoral. Toute modification de la loi Littoral doit être impérativement justifiée et encadrée, et les élus du littoral y sont extrêmement attentifs. Il ne s'agit pas « d'ouvrir la boîte de Pandore » en autorisant un « détricotage » de cette loi ; personne ne le souhaite. Ces dérogations à l'obligation d'urbanisation en continuité répondent à un besoin. Elles seront définies par les élus, les services de l'État et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre de stratégies de territoire, et se feront hors des espaces proches du rivage, à l'exception, bien entendu, cher Michel Vaspart, des cultures marines, qui nécessitent la proximité de l'eau.

Merci

et de s'adapter au phénomène de recul du trait de côte ». C'est cet impératif que rappelait Pascale Got, députée de la Gironde, dans sa proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Le texte que nous étudions cet après-midi- cela a été rappelé, mais je veux malgré tout insister sur ce point -reprend en quasi-totalité les dispositions défendues par ma collègue girondine il y a tout juste un an.

Une occasion manquée, donc, pour des dispositions qui proposaient, en plus de ceux existant déjà, des outils nouveaux à destination des communes, afin de mieux protéger les écosystèmes, d'aider à la gestion des zones soumises à l'érosion côtière, de sécuriser et d'harmoniser les documents d'urbanisme proposés par les élus et, enfin, d'apporter une solution à l'indemnisation des copropriétaires du Signal. Le volet préventif, prospectif, d'anticipation du texte est bien évidemment primordial,

Situé sur la falaise dunaire, construit il y a près de cinquante ans, dans le cadre des projets d'aménagement de la côte aquitaine, à l'origine à 200 mètres du front de mer, il a bénéficié d'un permis de construire accordé par l'État. Il est aujourd'hui face à un danger imminent d'effondrement. C'est ainsi que, dès 2011, les 75 propriétaires ont reçu un ordre d'évacuation définitive avec interdiction d'habiter ou de pénétrer dans les lieux, et ce sans indemnités, car ils seraient prétendument non éligibles au fonds Barnier. affaire a donné lieu, depuis lors, à une bataille juridique, bataille non aboutie à ce jour, puisque, sur décision du Conseil d'État, le dossier vient d'être porté devant le Conseil constitutionnel, qui va devoir se prononcer. Depuis la tempête de 2010, la situation de cette résidence fait périodiquement l'objet de nombreuses chroniques dans les médias, photos à l'appui. Ce qui n'est pas périodique, hélas ! c'est la situation intenable des propriétaires, pour la plupart de modestes retraités, expropriés, privés de leurs biens, contraints de se reloger à leurs frais. L'article 3 du présent texte crée un montage spécifique pour la mise en oeuvre d'un régime d'indemnisation transitoire. Celui-ci s'appliquerait pour les interdictions définitives d'habitation ou d'occupation des lieux résultant d'un risque de recul du trait de côte, lorsque des permis de construire auront été délivrés par les services de l'État. Le problème spécifique de l'indemnisation des copropriétaires du Signal, à Soulac-sur-Mer, trouverait alors une réponse, sans pour autant qu'un « effet d'aubaine » soit suscité. Ce ne serait que réparation. C'est pourquoi

Ce texte a notamment pour ambition de faciliter le recul stratégique des activités et le développement équilibré des territoires littoraux. Il s'inspire d'une partie des propositions du rapport sur l'application de la loi Littoral que j'avais rédigé, en 2013, avec notre collègue Odette Herviaux. Je me félicite d'y trouver des dispositions autorisant la densification des hameaux par comblement des « dents creuses », qui permettent la relocalisation des biens menacés par l'érosion littorale et les dérogations relatives aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines. Je rappelle tout de même, à l'attention de celles et ceux qui s'inquiéteraient que l'on puisse ainsi porter atteinte à la loi Littoral, que de nombreux garde-fous sont prévus : ces dérogations ne sont possibles qu'en dehors des espaces proches du rivage, dans des zones identifiées identifiées par un SCOT et délimitées par un PLU, et sont soumises à accord de l'administration, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites- autant de clés de sécurité. Au-delà de ces questions d'urbanisme, les territoires littoraux sont de plus en plus violemment confrontés aux effets du changement climatique, avec d'importants dégâts sur nos côtes, ce qui préoccupe les élus quant à la sécurité des personnes et la préservation des biens. Les réponses à apporter sont complexes, entre renforcement des ouvrages de défense contre la mer et reculs stratégiques. Chaque situation est particulière. En même temps, les aménagements réalisés par une commune peuvent avoir des conséquences sur le littoral des communes voisines. La stratégie de gestion intégrée du trait de côte est donc indispensable. À cet égard, je me félicite de la place que ce texte laisse aux initiatives locales. Mais, au-delà des outils juridiques, les élus sont bien souvent désemparés devant l'ampleur des travaux à réaliser. Nous devons donc les aider à supporter la charge financière que ceux-ci représentent. Je défendrai dans la suite de la discussion un amendement en ce sens. Il serait tout à l'honneur de la Haute Assemblée de voter un tel dispositif, que de nombreux élus locaux appellent de leurs voeux.

fait pour mettre en application les dispositions de la loi Littoral, si ce n'est, en 1989, un décret et une circulaire, qui ont plutôt complexifié la mise en oeuvre de la loi. Même si, depuis, d'autres textes ont été produits,

à la volonté du législateur. Depuis quelques années, le Sénat a eu à coeur de faire preuve de pragmatisme et d'ouverture par rapport à la loi Littoral.

qui seront nécessaires. Je ne saurais imaginer que votre ligne de conduite soit de laisser la nature faire les choses, sans pouvoir réagir. La

Les outre-mer, dont je suis l'un des représentants dans cet hémicycle, sont particulièrement concernés par la question des territoires littoraux et des facteurs de leur développement. En effet, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion comptent, à elles seules, 92 communes littorales. Plus grande île volcanique de l'archipel des Petites Antilles, la Martinique, la Martinique, qui compte environ 380 000 habitants, est la quatrième région française la plus densément peuplée, avec 344 habitants par kilomètre carré. Elle couvre 1 080 kilomètres carrés et est soumise à de nombreux risques naturels : séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, cyclones tropicaux, érosion côtière et glissements de terrain. La Martinique est ainsi, avec la Guadeloupe, le territoire français le plus exposé au risque sismique. Ayant été maire de la commune du François pendant de nombreuses années, je mesure parfaitement les enjeux et les difficultés propres à la thématique du développement durable des collectivités territoriales. si le recul du trait de côte est un phénomène auquel citoyens et pouvoirs publics se confrontent et se confronteront de plus en plus en raison du changement climatique, les conséquences humaines, matérielles, économiques et environnementales se font déjà sentir. Pourtant, il est difficile de se projeter et de se rendre compte de l'ampleur du phénomène à venir. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les communes du littoral constituent des lieux de contact et d'échanges très importants, qui abritent, par ailleurs, des milieux parmi les plus riches et les plus productifs de la planète. contribue fortement à l'attractivité de ces communes et de certains territoires pourtant exigus, comme la Martinique, ce qui crée des emplois et favorise l'économie, par le biais du secteur touristique. C'est pourquoi il est nécessaire de de trouver le juste équilibre entre urbanisme contrôlé et protection du littoral, tout en gardant en mémoire que certains territoires comme la Martinique manquent cruellement de foncier. Dans cet esprit,

La diffusion d'une culture du risque a également pour but de protéger les élus locaux, qui sont souvent confrontés à l'incompréhension de leurs concitoyens lorsque des mesures d'envergure doivent être prises. qu'élu de la côte basque, plus particulièrement de Biarritz, j'ai pu observer l'incompréhension des administrés confrontés à des procédures d'expropriation. Par manque de connaissance des risques, ces décisions sont mal comprises par les populations. Les élus locaux doivent parfois engager un véritable bras de fer, alors qu'ils agissent par devoir de prévention et par souci de sécurité de leurs concitoyens. Les exemples de ce type sont malheureusement nombreux. Ces expériences vécues par les élus locaux appellent notre attention et notre action. C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise que les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, élaborées par les collectivités ou leurs groupements, aient également pour mission de sensibiliser et de responsabiliser les citoyens à la fragilité de leur environnement et aux risques inhérents à celui-ci, en comportant des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Cet amendement tend à ce que les stratégies locales de gestion intégrée comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte.

Je partage le souhait de développer cette culture et cette mémoire du risque dans les territoires exposés au recul du trait de côte, mais, en l'état actuel de l'article 1, deux faiblesses sont à relever. Premièrement, les stratégies locales sont facultatives. Deuxièmement, leur contenu mériterait d'être revu plus largement, afin notamment de prévoir qu'elles puissent proposer la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement.

de manière très furtive concernant le fonds Barnier -un important problème de financement pour les collectivités, puisque ce ne sont pas les départements, les régions, les communautés d'agglomération ou les communes qui pourront faire face à ces choix douloureux et à ces coûts financiers. La

Consigne a été donnée aux services en ce sens une circulaire, et bientôt un arrêté. Il est préférable de conserver la fixation de ce niveau dans un document que l'on peut réviser rapidement et à tout moment, chaque fois que l'évolution des connaissances le nécessitera, plutôt qu'au sein du Plan national d'adaptation au changement climatique, dont la révision suit une procédure complexe et

Ce nouveau zonage doit permettre le maintien de constructions ou d'ouvrages pendant une durée déterminée dans des zones qui ne sont pas menacées de manière imminente par un risque de recul du trait de côte. Ces constructions peuvent alors être soumises à des prescriptions particulières. Ce nouveau zonage, qui avait fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de Pascale Got, est utile pour permettre de concilier le maintien des activités littorales et la prise en compte du risque de recul du trait de côte. La solution proposée par l'auteur

la solution la plus adaptée. Les outils d'aménagement, qui sont aux mains des collectivités, nous semblent plus adaptés à la réalisation de leurs projets de territoire en favorisant à la fois le développement économique et l'adaptation

elle en occulte sa spécificité due à la montée du niveau de la mer et à l'évolution des courants de marée et de houle. Les auteurs de cet amendement rédactionnel ont donc pour simple ambition de renforcer l'existence de ce risque dans les textes.

porte sur l'introduction des zones d'activités spécifiques à l'érosion dans les PPRN. Nous sommes défavorables à cet article, qui traite l'érosion des outils de politique des risques, ce qui nous paraît inadapté.

sorte de zone tampon où la collectivité se doterait des moyens de procéder à une évacuation progressive et à la relocalisation des activités. Si nous partageons l'idée d'anticipation et de préparation longue, nous ne souhaitons en aucune manière que ce nouveau zonage participe à l'urbanisation d'espaces pour lesquels le risque de submersion est avéré, seul le rythme étant sujet à aléa.

Or nous considérons que ne pas vouloir aggraver ce risque revient à interdire tout type de construction sur ce périmètre, et ce même de manière transitoire. Comme nous l'avons indiqué lors de la discussion générale, l'intérêt de ce texte réside dans l'adaptation des territoires littoraux aux phénomènes climatiques. Il n'a pas vocation à accroître les possibilités de construction.

Si une construction peut être autorisée de manière temporaire dans une zone d'adaptation au recul du trait de côte, il ne faut pas pour autant oublier la nécessaire prise en compte prise en compte des autres risques- notamment la submersion marine -pouvant justifier le caractère inconstructible de ladite zone. Ces constructions ne doivent donc pas être autorisées dans une zone rouge du PPR.

pour présenter l'amendement n° 25 rectifié. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de délimiter des zones de mobilité du trait de côte, les ZMTC, que j'ai évoquées lors de la discussion générale, dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

reprises que les PPRNP peuvent d'ores et déjà délimiter des zones rouges au sein desquelles des interdictions peuvent être mises en place. En conséquence, il n'estime pas nécessaire de prévoir un nouveau zonage.

où une protection spécifique de la biodiversité doit être mise en place. En effet, les zones rouges ne concernent que l'interdiction de construction, sans prendre en considération la vulnérabilité naturelle des écosystèmes. À l'inverse, le rôle de la ZMTC consisterait à définir un périmètre spécifique de protection des écosystèmes. écosystèmes. Une différence d'interprétation sur la portée de ce dispositif demeure. En commission, nous avons déposé cet amendement en demandant des explications que nous n'avons pas obtenues. raison pour laquelle, face à ces divergences d'analyse persistantes et aux risques que présenterait l'adoption d'un dispositif mal adapté à certaines réalités ou à certains territoires, nous souhaitons réintroduire la possibilité de délimiter des ZMTC.

pour présenter l'amendement n° 33. Le présent article modifie les zonages au sein des plans de prévention des risques naturels. Il permet ainsi, à la demande des collectivités territoriales, la création d'une nouvelle zone intermédiaire, transitoire et résiliente, afin de faire face spécifiquement au recul du trait de côte. Cette nouvelle zone serait ainsi créée à côté des zones de danger, dites zones rouges, dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées sous certaines conditions, voire interdites, et des zones bleues, qui ne sont pas directement exposées aux risques. La proposition de loi initialement débattue par la Sénat, en janvier dernier, instaurait une autre zone, dite « mobilité du trait de côte », dans laquelle les constructions, ouvrages et aménagements seraient purement et simplement interdits à l'exception des ouvrages de défense contre la mer, afin de permettre aux écosystèmes côtiers de s'adapter. En commission, le Sénat avait supprimé cette disposition au motif qu'il s'agissait d'un élément redondant par rapport aux zones rouges des PPRN, qui peuvent déjà comporter des mesures d'interdiction des constructions existantes ou futures, ainsi que des mesures d'autorisation assorties de certaines prescriptions. Nous ne partageons pas cette analyse : en zone rouge, les interdictions sont facultatives et ne couvrent pas l'ensemble de ladite zone. Un zonage spécifique d'interdiction de toute construction aurait l'avantage de la clarté. Par ailleurs, selon un certain nombre d'acteurs, et notamment le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, la biodiversité des territoires ultramarins nécessite une protection spécifique qui ne serait pas suffisamment prise en considération dans un simple zonage rouge.

tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales

ces amendements proposent la création de zones de mobilité du trait de côte dans les PPR afin d'interdire les constructions dans les zones soumises à l'érosion. La création de ces zones n'est pas nécessaire. correspondent en effet à une zone rouge classique d'un PPR, où sont interdites les constructions en raison de la présence d'un risque important. Je comprends que ces amendements visent à permettre, dans ces zones, la construction de digues ou d'aménagements pour la culture marine, mais il est déjà possible, dans les zones rouges d'un PPR, d'autoriser certaines constructions présentant des caractéristiques spécifiques. Les textes actuels répondent donc déjà au besoin soulevé ici.

il est urgent de trouver une solution pour aménager la loi Littoral sans renier son esprit ni sa nécessité. Cette loi ne peut-être un totem à tout jamais figé offrant au préfet non élu une trop grande liberté d'appréciation dont il use de manière parfois trop tatillonne. Nous ne pouvons passer d'un extrême à l'autre, de la « bétonisation » à tous crins au refus de tout microprojet temporaire ou saisonnier. La bande des 100 mètres, par exemple, empêche les campings municipaux de toutes petites communes de vivre, à la belle saison, comme à Taller, en Médoc.

Comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement est défavorable au principe qui consiste à traiter l'érosion des outils de politique des risques. Cela nous apparaît fondamentalement inadapté.

Il s'agit une nouvelle fois de rétablir dans cette proposition de loi un dispositif qui y figurait initialement. Ainsi, en janvier dernier, la commission et le rapporteur avaient choisi de supprimer la disposition concernant le droit d'information des acquéreurs et les obligations des agents immobiliers. L'ancien article 8 visait à imposer aux professionnels de l'immobilier d'informer les preneurs de biens du risque de recul du trait de côte lorsque les biens concernés sont situés dans une zone d'activité résiliente et temporaire. Ces professionnels sont aujourd'hui tenus d'un simple devoir de conseil, reconnu par la jurisprudence. Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant qu'elle était couverte par ce même devoir de conseil. Or le juge judiciaire ne l'entend pas ainsi, comme en témoigne l'arrêt du 10 février 2016 de la cour d'appel de Bastia, qui rappelle que « la responsabilité de l'agent immobilier

Il s'agit d'un élément de confiance pour le marché immobilier et d'une information primordiale pour les acquéreurs du bien, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Il ne s'agit pas, en outre, d'une obligation déraisonnable pour la profession.

lieu de l'acquisition. Dès lors, leur responsabilité est engagée sur le plan civil lorsqu'ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu'ils ignorent un vice caché. Par ailleurs, les informations relatives aux risques naturels sont d'ores et déjà présentes dans les dossiers de diagnostic technique annexés à la promesse de vente ou au bail de location.

Mme Corinne Imbert, sur l'article. L'article 9 vise à étendre les dérogations au principe d'extension en continuité de l'urbanisation dans les parties rétro-littorales des communes. Actuellement, ces dérogations sont limitées aux seuls terrains de camping, aires de stationnement de caravanes, activités agricoles et forestières et parcs éoliens. le cadre de la législation actuelle, certaines communes sont confrontées à des difficultés pour obtenir les autorisations d'agrandissement de campings existants. Pour autant, il ne s'agit pas de remettre en cause la loi Littoral de 1986. Je prendrai pour exemple la Charente-Maritime,

L'article 9 de la proposition de loi entend remédier à cette situation en rationalisant la question des dents creuses et des annexes ainsi qu'en cherchant des solutions pour les biens menacés par l'érosion.

le logement des travailleurs saisonniers. Il vise à créer un cas de dérogation relatif aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines mentionnant expressément le logement des saisonniers et du chef d'exploitation.

Comme l'a dit notre rapporteur en commission, il faudra reposer la question en séance, car les professionnels attendent des réponses concrètes et un cadre juridique protecteur. Tel est l'objet de ma démarche. Le texte ici proposé est plus équilibré que la version adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour l'article 9 Cette version permet de limiter à la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l'urbanisation, s'agissant de constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause

La constructibilité est strictement encadrée, contrairement à la version actuelle de cet article de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2017. En effet, sur le plan géographique, ne sont visés que les secteurs rétro-littoraux, situés en dehors de la bande des 100 mètres et en dehors des espaces proches du rivage, et non pas la totalité des territoires des communes littorales. Sur le plan économique, le logement des agriculteurs et de leurs salariés saisonniers est expressément autorisé sur les exploitations agricoles qui ont besoin d'une main-d'oeuvre durant les périodes de récoltes, la mention étant indispensable pour répondre à un besoin réel et faciliter la réglementation dans les documents locaux d'urbanisme et la délivrance des autorisations d'urbanisme. Sur le plan administratif, cette possibilité est conditionnée par la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que par l'obtention de l'accord préalable du représentant de l'État dans le département en tant que garant du respect de la loi Littoral.

nous avons pu le mesurer dans le cadre des différentes interventions à l'occasion de la discussion générale, nous sommes tous très attachés à la loi Littoral. Toutefois, si nous sommes ici aujourd'hui, sur l'initiative de Michel Vaspart et, avant lui,

la loi de 1986. Ces dernières années, elle n'a pas permis une approche équilibrée entre protection de l'environnement et développement local dans certains territoires. Je le rappelle, l'esprit même du développement durable, c'est de

savez tous ici, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement considère que les réflexions sur l'adaptation des territoires littoraux

de trente ans, à la protection des espaces naturels littoraux et à la lutte contre leur artificialisation. Elle constitue selon nous, avec les mécanismes de protection des espaces fragiles, un levier d'adaptation aux processus d'érosion. Bien sûr,

Repousser encore et encore la réflexion, les décisions ou l'évolution législative me semble non pas une erreur, mais une faute.

l'émergence et la concrétisation d'un certain nombre de projets de bon sens sur le littoral. Par conséquent, si on veut le développement équilibré de notre pays, il faut aussi que, dans les communes littorales, on puisse enfin construire de façon normale, sans qu'il s'agisse d'une urbanisation outrageante et d'une artificialisation outrancière de nos territoires. Le bon sens, comme vient de l'exposer très clairement Michel Vaspart, c'est de permettre, dans les dents creuses, c'est-à-dire dans les zones déjà construites, une densification.

l'identification, dans les schémas de cohérence territoriale, et la délimitation, dans les plans locaux d'urbanisme, des dents creuses pouvant être considérées comme

Je voudrais que nous affirmions ici, clairement et nettement, notre prise de conscience de la question du recul du trait de côte, mais aussi la nécessité de défendre nos littoraux par des aménagements intelligents. Il n'y a rien de mieux, en définitive, pour défendre nos

d'habitations dans les hameaux du littoral pose un vrai problème, que nous connaissons dans certaines régions, en particulier sur le littoral breton. Il se trouve que la Bretagne se caractérise par un habitat

aujourd'hui, c'est que nous sommes responsables de ce changement climatique. Il me semble donc complètement inutile d'avancer l'argument historique

l'évolution proposée, au travers de cette proposition de loi, par notre collègue Michel Vaspart, du droit à l'initiative et au bon sens des élus locaux ; mais pas pour faire n'importe quoi ! Certains ont fait des erreurs-

cette proposition de loi- et ce n'est pas la première fois que le Sénat se penche sur cette question -, donner plus de responsabilités et d'attention aux élus locaux.

est de tenter d'y répondre. L'article 9 vise à revenir sur le principe de continuité défini par le code de l'urbanisme. Sous couvert de répondre à une problématique spécifique, celle de permettre l'urbanisation des dents creuses, cet article ouvre une brèche immense dans les principes fondateurs de la loi Littoral. Certes, les dérogations prévues sont soumises à l'accord du préfet, mais nous connaissons tous les difficultés des préfectures, aujourd'hui, dans leur rôle d'accompagnement des collectivités locales. Nous craignons, à ce titre, un Il s'agit donc bien de contourner la jurisprudence constante des tribunaux, qui considère presque toujours les hameaux comme de l'urbanisation diffuse, au regard d'un faisceau de critères : l'accès au réseau, la densité, la qualité du bâti et la présence de services publics. Nous proposons, pour notre part, une autre démarche pour répondre à cette problématique. En premier lieu, nous proposons de supprimer la notion de « hameaux nouveaux », qui ouvre de nouveaux foyers d'urbanisation, à rebours des objectifs poursuivis, la loi Littoral, de lutte contre l'étalement urbain. C'est ce qui différencie d'ailleurs notre amendement de ceux déposés par d'autres groupes. Nous préférons en effet la densification encadrée et limitée au mitage du territoire. lieu, nous proposons de reconnaître légalement ces hameaux comme « des secteurs comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération ». Afin d'y permettre le comblement des dents creuses, nous posons deux critères : le nombre de constructions et leur distance les unes par rapport aux autres. Il s'agit de rapprocher ces critères de ceux utilisés pour l'application de la loi Montagne pour la définition d'un groupement. Enfin, en troisième lieu, nous proposons que ce travail de clarification s'incarne dans un décret en Conseil d'État, qui définirait très précisément toutes ces notions dont dépend la possibilité d'urbanisation. Il convient, en tout état de cause, d'être extrêmement prudent sur le sujet et de s'en tenir à la stricte problématique des dents creuses, c'est-à-dire du comblement d'une parcelle entre deux parcelles déjà bâties. Tout autre élargissement des possibilités de construction en discontinuité, que ce soit pour des installations agricoles ou pour relocaliser les anciens occupants des ZART,

ce que cet article a vocation à éviter. Elle supprime les autres dérogations relatives à la relocalisation dans le cadre des ZART aux constructions et installations liées à certaines activités et aux annexes.

Mais, compte tenu de la position de principe du Gouvernement sur cet article, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Je tiens aussi à dire que le Gouvernement n'est pas opposé par principe à toute discussion sur la loi Littoral. Nous sommes ouverts ouverts à des interprétations de clarification réglementaire de la loi Littoral. S'agissant de cette proposition de loi précise, elle traite de la question

nous n'envisageons aucune extension de l'urbanisation. Nous sommes contre l'extension de l'urbanisation ! Exactement ! Il faut vraiment prendre

moi, je suis très attaché à la loi Littoral ; c'est pourquoi je veux l'améliorer ! Je suis donc défavorable à cet amendement, mais il a au moins un mérite : en creux, ou en relief, je ne sais comment dire, il nous permet de défendre notre position en montrant que nous sommes si bien attachés, nous aussi, à la loi Littoral que nous ne voulons pas d'extension de l'urbanisation. Je crois l'avoir démontré.

en veillant toutefois à ce que la densification respecte des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l'installation de bâtiments volumineux.

savons pas très bien si elle est plus ou moins restrictive au regard de l'urbanisation diffuse existante. En tout état de cause, les élus locaux seraient alors libres de les identifier dans le cadre d'un PLU sans garde-fou autre qu'un règlement. La portée de cet amendement

Nous proposons de revenir à la rédaction de compromis qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale en seconde lecture lors de l'examen de la proposition de loi socialiste. Il convient ainsi de préciser, d'une part, que l'extension ne pourra avoir lieu que dans les hameaux existants et, d'autre part, qu'elle ne pourra être envisageable que dans des zones comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs, la définition de ce dernier critère étant renvoyée à un décret en Conseil d'État. Il s'agit d'encadrer le champ de la dérogation, afin d'éviter les effets d'aubaine et un risque de détournement de la loi Littoral. Si une construction totalement isolée venait à permettre une densification, nous remettrions en cause les fondements de cette loi. Nous sommes nombreux, au groupe socialiste du Sénat, à être très attachés à la loi Littoral, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des côtes relativement préservées. Les exemples malheureux de certains de nos voisins européens n'ayant pas réglementé leur urbanisation sur le littoral devraient nous inciter à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance en la matière.

Antiste. Afin de distinguer parfaitement le hameau du village, il importe au législateur d'en donner une définition au moins sommaire en reprenant celle qui a été donnée par le Conseil d'État à propos du hameau nouveau intégré dans l'environnement.

Son adoption restreindrait significativement la possibilité créée par l'article 9, en reprenant pour l'essentiel les critères consacrés par la jurisprudence en 2015- nous l'avons évoqué tout à l'heure

jugeant en particulier le critère de « faible importance » trop vague, donc sujet à des interprétations variables, sources de complexité et d'insécurité pour les acteurs locaux.

Cet amendement vise ainsi à préciser que les dérogations applicables aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines doivent être « nécessaires » à celles-ci, ainsi qu'à leur valorisation locale. En effet, la rédaction actuelle semble trop large en permettant toute forme d'extension dès lors qu'elle serait liée à une activité agricole, forestière ou marine. Nous avions présenté un amendement similaire en commission, mais il n'a pas été adopté. Toutefois, après des échanges avec M. le rapporteur, nous avons trouvé une rédaction de compromis ; le présent amendement en est la traduction.

des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées. Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue sous conditions aux éoliennes et à des stations d'épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux cultures marines, à des activités économiques et aux services publics d'intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation

des espaces. L'imprécision relative à la notion de services publics d'intérêt général et la généralité de la référence aux activités économiques nous inquiètent. Nous nous rapprochons de ce qui avait été un temps envisagé lors de la précédente proposition de loi

: La parole est à Mme Nelly Tocqueville. Toujours dans un souci de préservation de la loi Littoral, cet amendement vise à supprimer la dérogation que le présent texte entend accorder pour les édifications d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant. Si la rédaction actuelle de l'article encadre cette dérogation par un accord du préfet après avis de la CDNPS, il semble néanmoins que sa portée pourrait venir remettre en cause l'un des fondements de la loi Littoral en permettant des constructions en discontinuité de l'existant. Au-delà du fond, nous estimons qu'une telle dérogation ne doit pas être introduite dans le présent texte et qu'elle devrait faire l'objet d'une étude d'impact sur ses éventuelles conséquences et, de préférence, d'une proposition de loi à part entière.

dans la mesure où il ne doit pas simplement s'agir d'une construction qui existe en fait ; elle doit aussi être une construction légalement édifiée.

Quel est l'avis de la commission ? L'amendement n° 28 rectifié vise à supprimer la dérogation bénéficiant aux annexes de taille limitée à proximité des bâtiments existants. Cette dérogation reprend une disposition adoptée de manière consensuelle par les deux assemblées dans le cadre de la loi Montagne de décembre 2016. Il s'agit par ailleurs d'une demande ancienne des élus du littoral ; elle me semble suffisamment encadrée par l'ensemble des conditions de l'article que j'ai déjà évoquées. En visant des constructions de taille limitée et en renvoyant à la voie réglementaire pour préciser ces possibilités, nous avons une solution qui comporte des garanties supplémentaires.

On ne peut qu'être d'accord sur le principe, mais la faculté de vérifier une telle condition me semble délicate, d'autant plus que certaines procédures de régularisation existent, auquel cas il me semble complexe de revenir aux conditions initiales d'édification. Il appartient aux autorités locales

L'atteinte de ces objectifs implique une mobilisation des ressources disponibles sur l'ensemble du territoire national, qu'il soit urbain, rural, de montagne ou littoral. Or les équipements de production d'énergie renouvelable, en particulier les centrales thermiques solaires ou photovoltaïques photovoltaïques au sol, sont considérés comme des équipements urbains au titre de la loi Littoral. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme impose que les extensions d'urbanisation doivent se réaliser en continuité avec les zones agglomérées. Cette disposition contraint fortement le développement de projets de centrales de production énergétique, car les projets viennent potentiellement en concurrence avec la préservation des terres agricoles- prioritaire -ou avec l'accueil de nouvelles constructions. L'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance du 23 septembre 2015, permet aux projets d'implantation d'éoliennes de déroger au principe d'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbaines, sous certaines conditions. Le présent amendement vise donc d'élargir les dispositions de l'article L. 121-12 applicables à l'éolien aux centrales solaires, afin de permettre leur implantation en discontinuité d'urbanisation, notamment sur des espaces artificialisés par l'homme, tels que d'anciennes décharges réhabilitées, d'anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés. Cette proposition d'élargissement aux centrales solaires nécessite cependant une adaptation

par cet amendement, au développement des projets de centrales solaires sur l'ensemble de l'espace terrestre, y compris sur les communes littorales, est indispensable pour répondre aux enjeux de transition énergétique souhaitée par la population et pour favoriser le développement de l'autoconsommation collective, dont les modalités ont été définies par la loi.

L'objet de cet amendement est identique à celui de mon collègue Joël Labbé,

plus mesurée, qui répond à notre souci de ne pas trop étendre leur implantation en discontinuité de l'urbanisation existante et de la confiner à un certain nombre d'espaces bien identifiés. À l'heure actuelle, sur le plan national, environ sept dossiers sont bloqués

sur l'amendement n° 40. L'étalement tout au long de l'année de la fréquentation des zones littorales soulève un certain nombre de défis pour les communes qui doivent continuer d'assumer des missions de police des baignades et d'assistance en dehors des périodes estivales. Dans le même temps, ces mêmes collectivités font face à une diminution de leurs ressources. Ainsi, elles font de plus en plus appel à des associations de sauveteurs et de secouristes volontaires, qui assurent ces missions en dehors des périodes estivales ou en renfort pendant les pics de fréquentation. Intervenant de manière ponctuelle et en appui de la commune, les associations ne sont pas toujours reconnues comme un service public ni comme étant délégataires d'une mission de service public. L'article L. 121-17 du code de l'urbanisme dispose que l'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics. Cette disposition n'empêche pas que des communes aient des difficultés à procéder à des aménagements légers pérennes, comme des locaux de stockage du matériel, des vestiaires ou des douches pour ces associations. demeurent ainsi accueillies dans des bâtiments modulaires, dont l'insertion dans l'environnement est discutable, alors que dans les faits elles exercent une mission de service public. Cette situation spécifique est, par exemple, rencontrée dans mon département par la commune d'Anglet, dont le permis de construire a été contesté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif. Le permis a donc été annulé, ce qui a contraint la ville d'Anglet à conserver des bâtiments modulaires. Ainsi, je propose d'étendre de manière explicite l'exception d'inconstructibilité dans la bande des 100 mètres aux constructions nécessaires à l'exercice des missions de surveillance des plages, de secours et mer et de sauvetage côtier.

et empêcher, à terme, toute construction nécessaire aux exploitations agricoles ou conchylicoles. L'article 9 vise à interdire expressément les changements de destination de ces constructions, ce qui devrait permettre d'éviter ces dérives. À l'inverse, en interdisant toute habitation, on s'écarterait de la jurisprudence existante, qui autorise dans certains cas

la commission sur l'amendement n° 43 ? Cet amendement vise à ajouter aux dérogations prévues dans la bande littorale les constructions ou installations nécessaires aux missions de surveillance des plages, de secours en mer et de sauvetage côtier.

mesurer la nécessité d'une disposition législative. Modifier la législation sur le fondement d'un cas d'espèce n'est pas une pratique particulièrement favorable à la qualité de la loi. Il serait

? Quel est l'avis du Gouvernement ? La multiplication dans la loi elle-même de dispositions visant à résoudre des situations très particulières est contraire à l'esprit de la loi Littoral et n'est pas dénuée de risques contentieux des raisonnements. Un avis Un avis défavorable est d'autant plus justifié que de tels équipements semblent déjà couverts par les dispositions actuelles.

Ce besoin est particulièrement prégnant sur des territoires pour lesquels les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet amendement vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d'une main-d'oeuvre durant les périodes de récoltes. Cette version permet de limiter à la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l'urbanisation s'agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement, dont la mention explicite est indispensable afin d'en faciliter la réglementation au niveau local. Je me permets de souligner que deux agriculteurs

Ce sujet avait déjà été évoqué lors de la précédente proposition de loi. Créer une dérogation spécifique sur ce point, avec des imprécisions sur certaines notions, notamment celle de maîtrise et d'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, me semble révéler qu'une telle disposition n'est pas de niveau législatif. Vous citiez le chiffre

fondateurs de la loi Littoral. En tout état de cause, l'objectif visé par cet amendement est déjà satisfait. En effet, il revient au SCOT et au PLU de planifier les capacités d'accueil, en particulier dans les communes littorales où le foncier est très contraint, et d'identifier les secteurs destinés à accueillir des logements pour les saisonniers agricoles dans le respect des dispositions de la loi Littoral. Les collectivités se sont d'ores et déjà saisies de la question à travers leurs documents de planification. À titre d'exemple, le SCOT du pays de l'Or prévoit des dispositions visant à faciliter l'accueil des travailleurs saisonniers dans le respect de la loi Littoral, à savoir une intégration prioritaire dans le tissu urbain et dans le tissu villageois local.

: La parole est à M. Guillaume Chevrollier. En cohérence avec l'objectif visant à en encourager le développement durable des territoires littoraux, le présent amendement a pour objet d'étendre aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire le dispositif applicable aux éoliennes, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lorsque l'implantation de ces installations est incompatible avec le principe général d'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées. Bien entendu, l'implantation de ces équipements devra se faire dans le respect des conditions prévues à cet article, c'est-à-dire en dehors des espaces proches du rivage et en veillant à ne pas porter atteinte à l'environnement, aux activités agricoles, ainsi qu'aux sites et aux paysages remarquables. Concrètement, l'objectif est de pouvoir utiliser des espaces déjà artificialisés, tels que d'anciennes décharges réhabilitées, d'anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés,

Les dispositions d'urbanisme prévoient que l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages. Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence et doivent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non. Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés- anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau -, ne peuvent aboutir, sont considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante. Le cahier des charges du 11 décembre 2017 de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire, photovoltaïque ou éolienne indique, pages 9 et 10 du document, les quatorze types de sites dégradés ou prioritaires sur lesquels l'implantation d'installations photovoltaïques peut être envisagée, sous réserve d'être en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Or on admettra aisément que les sites dégradés peuvent ne pas être en continuité de l'urbanisation. Dans l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, la communauté de communes est porteuse de trois projets, situés dans des zones dégradées. À ce jour, ils sont bloqués, alors qu'ils représentent 3 gigawatts de production électrique par an soit 10 % de l'objectif TEPOS, territoires à énergie positive, à horizon de 2030. Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour permettre l'autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale, à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

est à M. Christophe Priou. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit le principe selon lequel « l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement La création d'une installation de traitement ou de stockage de déchets est considérée par la jurisprudence comme une extension de l'urbanisation soumise à ce principe de continuité, selon le tribunal de Marseille. Les communes littorales sont donc soumises à un régime plus strict que celles soumises à la loi Montagne, qui admet une rupture de continuité avec les espaces urbanisés pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage. L'amendement proposé vise donc à harmoniser les dispositifs de la loi Littoral et celui de la loi Montagne et tend à aligner le régime juridique des installations de services publics de traitement ou de stockage de déchets avec celui des éoliennes, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l'environnement, ce qui permet ainsi de revaloriser utilement un site dégradé.

proches du rivage. Actuellement, l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme prévoit qu'une telle dérogation est possible s'agissant d'installations éoliennes, lorsque celles-ci ne peuvent être installées à proximité de zones habitées. Il paraît cohérent, tant au regard des ambitions de transition énergétique que de l'objectif de développement durable des territoires littoraux, d'autoriser la construction de centrales solaires sur d'anciens sites d'usines ou de décharges à l'arrêt, qui pourraient ainsi être réhabilités et valorisés. Actuellement, les appels d'offres lancés par le Gouvernement relatifs à la construction de centrales solaires prévoient explicitement, comme l'une des conditions possibles d'implantation, le fait de créer une installation solaire sur un site dégradé. Ces appels d'offres définissent d'ailleurs précisément la nature de ces sites : il peut s'agir d'un ancien site pollué, d'une ancienne installation de stockage de déchets, d'un ancien aérodrome ou d'une friche industrielle. D'autres sites sont également possibles.

; d'autre part, il n'est pas justifié s'agissant de projets photovoltaïques, qui, à la différence des projets éoliens, ne sont pas soumis à des distances d'éloignement.

fondateur de la loi Littoral, est inopportun de manière générale alors que le taux d'artificialisation des sols sur les communes littorales

ne définit pas la notion de site dégradé. Il ne définit pas non plus un équilibre clair, qui doit pourtant être trouvé, avec la loi Littoral.

montagne, un PLU. Nous sommes réticents à modifier de telles règles, sans connaissance préalable des effets de ces modifications. Diviser par deux la largeur de la bande littorale, qui vise précisément à faire prévaloir un principe d'inconstructibilité sur la partie la plus sensible du rivage, n'est pas sans conséquence pour le territoire,

savez tous ici, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement considère que les réflexions sur l'adaptation des territoires littoraux à l'érosion du trait de côte ne doivent pas être l'occasion de remettre en cause la loi Littoral, qui participe de la protection des espaces naturels littoraux et de la lutte contre l'artificialisation des sols depuis plus de trente ans. Cela a été rappelé, notamment par le sénateur Dantec,

un levier de plus d'adaptation au processus d'érosion. Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut être que défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur la protection des espaces naturels situés à proximité immédiate du rivage des grands lacs, au motif qu'ils seraient artificiels.

: La parole est à M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à atténuer certains freins au développement du numérique et du très haut débit sur tout le territoire, en encadrant, sans l'interdire par principe, l'atterrage de nouveaux câbles sous-marins sur les côtes françaises. Le dispositif proposé s'inscrit pleinement dans l'engagement gouvernemental de résorber la fracture numérique et, en particulier, dans la démarche portée par le secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires. En effet, en l'état actuel de la législation en matière d'urbanisme, aux abords de la bande littorale, des constructions ou installations nouvelles de câbles peuvent être interdites soit au titre de la protection légale des 100 mètres du littoral, soit au titre des espaces remarquables mis en place par une collectivité locale. Le présent amendement a pour objet d'harmoniser le traitement des ouvrages de communications électroniques avec celui des ouvrages électriques, nécessaires à l'exercice des missions de service public telles que définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Ces ouvrages de communications électroniques remplissent également des missions de service public et d'intérêt général comme définies à l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques. Ce faisant, il prévoit bien que ces installations fassent l'objet du même niveau d'exigence que les ouvrages électriques, à savoir qu'elles soient à la fois « souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental

Il s'agit de composantes essentielles aux réseaux à très haut débit. Partageant la priorité définie par le Gouvernement en faveur de l'aménagement numérique du territoire, ces ajustements nous semblent pertinents et d'autant plus justifiés qu'ils se rattachent, concordance bienvenue, à un régime existant pour l'électricité. J'ajoute qu'un tel dispositif présente de vraies garanties environnementales, puisque les articles visés exigent le recours à des techniques souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Par ailleurs, ces opérations sont précédées d'une enquête publique. La commission a donc émis un avis favorable

Le sujet mérite d'être approfondi, alors que la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques est une priorité du Gouvernement et que nous avons déjà beaucoup avancé en la matière. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Le patrimoine architectural situé dans les zones classées au titre des espaces et milieux remarquables participe pleinement et conjointement à la valorisation du littoral et des sites classés. Il s'agit donc de permettre un changement de destination de ces bâtis remarquables pour empêcher leur disparition par l'élaboration d'un projet touristique et économique nouveau. Cette valorisation doit se faire dans le respect et en harmonie avec le site et le projet de territoire définis par les communes.

ne doit pas obérer le développement durable de ces derniers. Il s'agit donc de permettre la valorisation des patrimoines locaux remarquables qui s'inscrivent dans le paysage tout en donnant les moyens à des projets locaux d'émerger ; je pense notamment à des projets touristiques venant en complément des activités agricoles. Ce changement de destination se ferait

En réalité, les changements de destination n'y sont pas interdits par principe. Il revient aux collectivités territoriales de préciser dans leurs documents d'urbanisme les règles relatives à ces changements selon les espaces considérés et de les appliquer dans le cadre des autorisations d'urbanisme. À ce titre, nous ne voyons pas bien l'intérêt d'un tel ajout, sauf à envisager un changement qui serait « de droit », auquel cas cela remettrait en cause les compétences d'urbanisme des collectivités territoriales.

en dépit des règles prises par le plan local d'urbanisme et de l'instruction des autorisations du droit des sols assurée par l'autorité compétente. Serait instauré par la loi un régime dérogatoire, qui priverait les collectivités locales de leurs compétences

Une telle modification aurait une portée considérable, car elle reviendrait à soustraire à la loi Littoral toutes les communes situées autour d'un lac d'une telle superficie, même en dehors de l'Aveyron ! Plusieurs lacs et étangs sortiraient de ce régime et perdraient les protections qui résultent de la loi,

mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement considère que les réflexions sur l'adaptation des territoires littoraux à l'érosion du trait de côte ne doivent pas être l'occasion de remettre en cause la loi Littoral, qui participe de la protection des espaces naturels

trouver des voies et des issues pour travailler main dans la main à défendre notre paysage, notre biodiversité, tout en adaptant la législation aux réalités locales. En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, une situation ponctuelle ne pouvant justifier une remise en cause de la loi Littoral.

En effet, de nombreux garde-fous sont prévus, comme la constitution d'une garantie financière ou la nécessité de l'accord préalable du bailleur pour certaines actions, et le preneur doit respecter ses obligations contractuelles, notamment celle de maintenir en bon état d'entretien les constructions

figurant à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel interdit toute atteinte à l'état naturel du rivage. Je partage, monsieur le sénateur, le diagnostic que vous avez posé sur l'importance de la gestion des ressources en sable pour lutter contre l'érosion côtière. Pour autant, il n'est pas utile de modifier cet article du code général de la propriété des personnes publiques pour autoriser une telle opération, la liste des dérogations étant rédigée de façon suffisamment ouverte pour que de nombreuses actions de remise en place ou de rechargement, sous réserve qu'elles ne modifient pas le profil de la plage, puissent être réalisées.